madame la présidente.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

n'est pas défendu.

Ainsi, entre 2011 et 2016, le nombre de centres dentaires a progressé de 25 %. Parallèlement à cet assouplissement, et paradoxalement, le nombre de contrôles a diminué. Des centres dentaires à vocation lucrative

Faire intervenir les ARS pour l'implantation de tout centre de santé dentaire ou ophtalmologique est disproportionné et complètement inégalitaire, dans la mesure où aucune mesure de réglementation n'est prévue pour le Enfin, et je n'ai malheureusement pas le temps de développer davantage, il semblerait que le dispositif mis en place, notamment la transmission des diplômes et contrats des professionnels, présente le risque d'être inopérant. L'amendement

amendement tend à renforcer la portée réputationnelle des sanctions financières susceptibles d'être prononcées par le directeur général de l'ARS à l'encontre des gestionnaires de centres de santé ne respectant pas la réglementation. Il est ainsi prévu de donner au directeur général la possibilité de mettre le gestionnaire en demeure de publier les décisions de sanction financière le concernant sur le site internet du centre de santé en cause lorsque ce site existe, ainsi que, le cas échéant, sur les plateformes de prise de rendez-vous médicaux. Si la commission a choisi de conserver et amender cet article, c'est qu'il a une portée financière, prévoyant des pénalités et sanctions financières.

Dans le contexte de crise économique que nous traversons, les fraudes sociales constituent une perte de ressources importante. La lutte contre la fraude aux prestations sociales doit être accentuée. Pour cela, les sanctions à l'encontre des fraudeurs doivent être plus dissuasives. L'objet du présent amendement est donc de renforcer les sanctions à l'égard des fraudeurs aux prestations sociales dont la volonté de tromper l'administration est établie, ou de personnes en état de récidive. Il prévoit que des procédures à l'égard de personnes à qui des faits se rapportant à une fraude aux prestations sociales sont reprochés ne peuvent pas être abandonnées et qu'en l'absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, une contrainte soit systématiquement délivrée et une majoration des pénalités de 20 % soit systématiquement appliquée.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a déjà porté le plafonnement de la sanction de 50 % à 70 % des sommes concernées. Par ailleurs, cet amendement tend à supprimer le pouvoir d'appréciation du directeur de l'organisme local d'assurance maladie en lui retirant la possibilité d'abandonner des poursuites. Quelle que soit l'importance des enjeux, il ne paraît pas souhaitable de lier les mains du détenteur du pouvoir de sanction et de verser dans le « systématisme » : le principe de proportionnalité doit rester applicable à ces sanctions. En outre, l'amendement vise à modifier un ancien article du code de la sécurité sociale, qui n'est plus en vigueur. Pour toutes ces raisons, l'avis est défavorable.

Meunier, pour présenter l'amendement n° 623 rectifié. Les centres de santé participent à la politique de maintien à domicile des personnes âgées et handicapées. Outils de prévention des hospitalisations, ils s'inscrivent pleinement dans la stratégie Ma santé 2022. Reconnus par le code de la santé, ces centres sont aussi une réponse à la désertification médicale, mais leur pérennité est menacée, leur situation financière de plus en plus précaire, et ils ne peuvent pas absorber les augmentations légitimées par le Ségur de la santé, et prévues à son la branche de l'aide à domicile, qui se matérialisera par une augmentation de 15 % en moyenne de la masse salariale. Dans mon département de la Loire-Atlantique, le centre de santé d'Ancenis emploie 17 infirmières. Le calcul est vite fait : l'évolution de la rémunération entraîne un surcoût de 90 000 euros. Si l'on estime que les fonds propres de l'organisation gestionnaire sont de 150 000 euros environ, l'espérance de vie de ce centre de santé ne dépassera pas deux à trois ans. ans. Dans quelques mois, si rien n'est envisagé, c'est l'ensemble des activités de ces centres qui sera en péril et qui devra s'arrêter, laissant ainsi encore un grand nombre de patients sans réponse.

Je rappelle que les centres de soins infirmiers facturent à l'acte : ils peuvent donc faire varier leur rémunération en adaptant leur activité et ainsi bénéficier des revalorisations décidées dans le cadre conventionnel.

le Défenseur des droits indiquait, à la suite d'une enquête menée dans ce cadre, que 47,3 % des Guadeloupéennes et des Guadeloupéens et 45 % des Martiniquaises et des Martiniquais citaient l'accès aux soins comme l'une de leurs priorités.

L'amendement n° 365 rectifié prévoit que l'expérimentation de l'accès direct aux masseurs-kinésithérapeutes devra être réalisée dans « au plus six départements d'une même région ». Il est vrai qu'une expérimentation conduite au niveau régional permettra de garantir une meilleure coordination de son déploiement sous l'égide de l'ARS.

de compétences ; on reste au coeur du métier. Par ailleurs, la rédaction proposée est de nature à rassurer le corps médical, puisque la prescription médicale sera toujours possible. De même, les comptes rendus de visite chez un orthophoniste devront être transmis au médecin. La Fédération nationale des orthophonistes estime que près de 20 % des prescriptions médicales de bilan orthophonique, que les orthophonistes sont réglementairement tenus de réaliser, ne sont pas nécessaires et relèvent d'un mauvais adressage, tout simplement parce que les médecins ne sont pas formés à ces questions. Favoriser l'accès direct peut y remédier en permettant une meilleure prise en charge des patients alors que l'on connaît les difficultés pour obtenir des rendez-vous chez un orthophoniste. Au-delà de cette question de l'accès direct, j'en profite, monsieur le secrétaire d'État, pour vous demander si vous comptez augmenter le quota de professionnels. Partout, le manque d'orthophonistes

l'avis de la commission

Cet amendement apporte plusieurs précisions afin de mieux encadrer l'expérimentation de l'accès direct aux orthophonistes. Le décret devra être pris en Conseil d'État après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Académie nationale de médecine. Il est rappelé que l'orthophoniste a accès au dossier médical partagé,

soit inclus dans l'expérimentation visant à permettre l'accès direct pour les patients aux soins pratiqués par les orthophonistes lorsque ces derniers exercent dans une structure d'exercice coordonné.

D'après les études qui y ont été consacrées, ces doses sont nettement sous-estimées, de même que les risques liés aux faibles doses de rayons X. Pourtant, la place des examens scannographiques dans la prise en charge du patient ne cesse de croître. Or le scanner est l'examen le plus irradiant en imagerie diagnostique. Un acte délivre une dose environ 100 fois supérieure à celle que délivre une radiographie conventionnelle. Cette irradiation n'est pas sans risque pour la population : il existe un excès statistiquement significatif de risque de cancer à partir d'une dose cumulée de 100 millisieverts chez l'homme. L'enfant est particulièrement exposé du fait de la radiosensibilité importante de ses organes. Depuis la directive européenne 97/43, les professionnels de santé sont dans l'obligation d'estimer les doses d'irradiation reçues par leurs patients afin d'améliorer le suivi de l'exposition de la population aux rayonnements ionisants. Cette information est consignée dans le compte rendu de chaque examen, mais il n'existe actuellement aucun suivi des doses de rayonnements reçues par un patient au long de sa vie. Le médecin généraliste doit pouvoir établir un suivi d'irradiation pour chacun de ses patients. s'inscrit dans son rôle en soins primaires, d'éducation de ses patients et de prévention des risques sanitaires. Pour mettre en place ce suivi, il conviendrait d'aller plus loin que l'accès des médecins déjà possible au guide des bonnes pratiques il faudrait inscrire dans le dossier médical partagé la dose efficace cumulée reçue par examen d'imagerie médicale utilisant les radiations ionisantes. article, inséré par l'Assemblée nationale, vise à expérimenter dans six départements le financement par le fonds d'intervention régional de la mise à disposition de l'accès gratuit, dans l'espace numérique des médecins généralistes, au guide du bon usage des examens d'imagerie médicale. L'accès au guide étant déjà gratuit- il est disponible sur le site de la Haute Autorité de santé -, cette mise à disposition ne paraît pas nécessiter autre chose qu'un renvoi vers son site internet au sein de l'espace numérique des médecins généralistes. En ce qui concerne la campagne d'information prévue par le présent article, son ciblage très particulier ne paraît pas justifier de moyens spécifiques. Par ailleurs, l'intérêt direct pour les généralistes de l'usage de ce guide ne semble pas nécessiter d'actions approfondies, au-delà de courriers qui peuvent leur être adressés. Enfin, de telles campagnes d'information ne sont pas du domaine de la loi. En conséquence, la commission souhaite

Cette possibilité de primo-prescription est donc indispensable. Par ailleurs, nous avons reçu de nombreuses demandes pour que cet article permette l'accès direct des patients aux IPA. Pourquoi ne pas l'avoir inclus dans votre amendement, monsieur le secrétaire

Je tiens à me faire l'écho du mouvement de fond qui agite nos hôpitaux, nos cliniques et nos établissements de santé en général. L'article 41 élargit les responsabilités des infirmiers en pratique avancée en leur permettant, sous la forme d'une expérimentation, de réaliser « certaines prescriptions soumises à prescription médicale dont la liste est fixée par décret ». Monsieur le secrétaire d'État, n'entendez-vous pas les IADE et les Ibode qui se mobilisent dans tout le pays ?

Où sont les engagements pris pour une vraie reconnaissance de la profession ? N'oubliez pas que, si les IADE se limitaient strictement à ce que permet leur statut, il n'y aurait plus d'anesthésies en France.

Afin de garantir la diversité des territoires investis dans ce dispositif ainsi que leur représentativité, cet amendement vise à garantir la présence d'une région ultramarine.

le constat était déjà inquiétant : l'obésité chez les enfants progresse en France. Mauvaises habitudes alimentaires, malbouffe, sédentarité accrue

généralise l'expérimentation des parcours de prise en charge de l'obésité : il faut saluer l'ambition et les bonnes intentions de cette mesure. Mais l'entrée dans ces parcours ne faisant l'objet d'aucune obligation, elle ne reposera que sur l'attention des parents à la santé de leur enfant.

puis une orientation vers les professionnels de santé auraient permis de toucher toute une classe d'âge à échéances précises, par exemple à 3, 6 et 12 ans. Nous le savons : en dehors de quelques villes, comme celle de Nantes, qui ont conservé un service municipal de santé scolaire, la médecine

(PMI). Les services de santé scolaire ont un rôle déterminant à jouer dans la prévention du surpoids et de l'obésité chez les enfants. Les médecins de l'éducation nationale et les médecins des services de PMI figurent parmi les principaux interlocuteurs des familles et des enfants en matière de prévention, pour les enfants les plus défavorisés sur le plan socioéconomique, qui ne sont pas nécessairement suivis par un médecin de famille. conséquence, cet amendement tend à préciser que les centres et maisons de santé mettent en oeuvre le parcours d'accompagnement des enfants en situation de surpoids, en collaboration avec le médecin de l'éducation nationale de l'établissement dans lequel est scolarisé l'enfant et, le cas échéant, avec le médecin traitant ou le médecin du service de PMI, bien sûr toujours avec l'accord des parents. Cet amendement vise également à inscrire parmi les missions des médecins de l'éducation nationale et des médecins des services de PMI la participation à la mise en oeuvre du parcours, afin de leur reconnaître la capacité d'orienter l'enfant et sa famille vers un centre de santé ou une maison de santé susceptible d'assurer cette prise en charge.

recueils et traitements de signaux biologiques à visée de dépistage, d'orientation diagnostique ou d'adaptation thérapeutique immédiate. Ces différents tests, recueils

La crise sanitaire l'a démontré : la stratégie de dépistage est efficace lorsque le patient peut accéder facilement à un test réalisé par un professionnel de santé ou une personne habilitée. Le patient peut ensuite être orienté plus rapidement vers un médecin et entrer éventuellement dans un parcours de soins adapté. est l'avis de la commission

par le fait que le mode de rémunération n'y est pas favorable. Actuellement, le modèle de financement de la radiothérapie est inadapté, car il repose sur un système de double tarification qui engendre des distorsions tarifaires et une mauvaise allocation des ressources. Ce constat, qui n'est pas nouveau, est dressé à la fois par les pouvoirs publics, l'assurance maladie, les professionnels de radiothérapie et les fédérations hospitalières. Une expérimentation d'une durée de quatre ans a été lancée en vertu de l'article 43 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014. Elle a permis de confirmer l'évolution vers un modèle de financement forfaitaire, mais la concrétisation de cette réforme se fait encore attendre. L'assurance maladie le souligne pourtant dans son rapport sur l'évolution des charges et des produits au titre de 2017 : cette réforme est nécessaire,

cet amendement tend à inscrire dans la loi l'aboutissement programmé de la réforme du financement de la radiothérapie, engagée il y a près de dix ans. Compte tenu des économies escomptées, cet aboutissement mérite d'être inscrit parmi les travaux prioritaires du Haut Conseil des nomenclatures

vers un modèle de financement forfaitaire, mais la concrétisation de cette réforme est toujours attendue. La commission des affaires sociales a déjà réclamé au Gouvernement la transmission du rapport d'évaluation de l'expérimentation de la forfaitisation du financement de la radiothérapie. Cependant, elle n'a obtenu aucune réponse, ni même un accusé de réception de sa demande. Le financement par forfait est mieux adapté à la prise en charge des techniques de radiothérapie innovantes, notamment la radiothérapie conformationnelle avec modulation d'intensité développée depuis 2010, qui permet une meilleure focalisation des rayonnements sur la tumeur.

objectifs : améliorer la prise en compte du parcours de soins du patient, mieux répondre aux enjeux de qualité et de sécurité des traitements, tenir davantage compte des évolutions technologiques et de l'innovation, mieux maîtriser l'évolution des dépenses dans les deux secteurs- hospitalier et libéral -, et enrichir le suivi et les connaissances sur le traitement du cancer par radiothérapie par la mise en place d'un recueil d'informations médicalisées adapté. Le périmètre envisagé jusqu'à présent pour le nouveau modèle inclut les localisations du sein et de la prostate.

effet, le « couperet » du tarif peut empêcher une population extrêmement captive de se rendre chez ces professionnels.

par un médecin généraliste retarderait considérablement la démarche de consultation psychologique, ce qui n'entraînerait pas forcément une économie pour l'assurance maladie. cela engendrerait plusieurs consultations médicales remboursées. Les psychologues sont des professionnels de santé mentale formés au niveau master 2 de l'université. Le dispositif proposé imposerait la durée et le nombre des consultations prévues, ce qui n'est pas adapté à la réalité De plus, la tarification très basse, à 30 euros, proposée par le Gouvernement, ne serait pas favorable au maintien d'un exercice libéral dans des conditions acceptables, en raison des nombreuses charges qui incombent aux psychologues.

sachant que chaque patient a une histoire différente ? Comment ignorer que la fixation d'un nombre préalable de séances est contraire à l'esprit d'une psychothérapie, qui doit être individualisée en fonction du patient ou de la patiente ? Notre deuxième point de désaccord a trait au tarif des consultations, qui est trop bas.

Compte tenu des besoins d'accès aux soins en santé mentale et de l'augmentation des risques psychosociaux associés au travail, la mise en place de séances d'accompagnement psychologique entièrement prises en charge

prise en charge de séances pour l'ensemble de la population souffrant de troubles psychiques- d'intensité légère à modérée -doit permettre d'améliorer l'accès aux soins en santé mentale. Il s'agit d'une mesure majeure pour améliorer la santé mentale de nos concitoyens.

entre le psychologue et le médecin

Les agences régionales de santé, qui arrêtent les projets territoriaux de santé mentale, sont les mieux placées pour sélectionner les psychologues participant au dispositif des séances d'accompagnement psychologique. Les deux amendements suivants sont identiques. L'amendement

Selon Santé publique France, 23 % des adultes déclarent des signes d'anxiété, soit dix points supplémentaires par rapport au niveau d'avant la crise. De plus, 10 % des Français ont eu des pensées suicidaires au cours de l'année, soit cinq points de plus d'avant la crise. Enfin, chez les enfants et les jeunes adultes, le nombre de passages aux urgences pour geste suicidaire a fortement augmenté. La santé mentale a été souvent, longtemps, la grande oubliée des politiques de santé. La crise sanitaire a révélé et démultiplié les manifestations

à un prix plafonné à 30 euros. Comment peut-on faire croire qu'une dizaine de séances suffira toujours pour accompagner un patient en souffrance ? En outre, que se passe-t-il à l'issue de ces séances ? Comment ignorer l'insuffisance de la rémunération au regard du temps moyen de la consultation, et la paupérisation de la profession qu'elle sous-tend ? Faute de pouvoir amender le dispositif sur ces points, je vous invite à retenir le présent amendement qui vise à intégrer les représentants de la profession de psychologue au sein de l'autorité sélectionnant les psychologues, afin d'enrichir les critères de sélection à partir de leurs pratiques et de leurs compétences.

les psychologues habilités à réaliser des séances d'accompagnement psychologique, l'amendement n 1001 tend, quant à lui, à confier cette sélection à une autorité composée uniquement de représentants de la profession de psychologue.

Plus globalement, la généralisation de la prise en charge de séances d'accompagnement prolonge une démarche qui reste expérimentale. Il sera probablement nécessaire d'ajuster les modalités de sélection au fur et à mesure de la mise en oeuvre-

Afin d'encourager une dynamique de coopération et de coordination entre les professionnels médicaux et les psychologues, l'amendement prévoit que le psychologue,

un adressage au psychologue par le médecin ayant repéré une situation de détresse psychologique. Il est donc nécessaire d'intégrer le psychologue dans l'équipe de soins. Cette intégration permet de lui appliquer l'exigence de partage d'informations strictement nécessaires à la coordination ou à la continuation

de même que les soins psychologiques sont importants sur le plan physique. Il y a une complémentarité entre la tête et les jambes, comme on

Comme le rappelait la ministre déléguée chargée de l'autonomie, Mme Brigitte Bourguignon, lors des discussions à l'Assemblée nationale, « cette mesure vise des patients souffrant de troubles dépressifs ou anxieux, d'intensité légère à modérée. Toute la population âgée d'au moins 3 ans peut en bénéficier ». Or il paraît opportun d'appliquer le principe de ce dispositif aux victimes de violences intrafamiliales. Celles-ci sont souvent confrontées à des barrières financières, à une prise en charge insuffisante dans le temps, ainsi qu'à la difficulté de trouver un professionnel pour les aider. Le dispositif prévu par ce texte, avec une prise en charge financière complète de huit séances pour les patients qui en ont besoin, semble

Un Français sur cinq est touché, chaque année, par un trouble psychique, soit 13 millions d'entre eux ; 64 % des Français ont déjà ressenti un trouble ou une souffrance psychique ; les Français sont les plus gros consommateurs au monde de psychotropes le suicide est la deuxième cause de mortalité entre 10 et 25 ans. Ces chiffres sont un appel à agir et nous nous félicitons de l'introduction de cet article dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, qui permettra de soutenir concrètement la santé mentale des Français. Dans ce cadre, cet amendement vise à assurer que la répartition des psychologues prenne en considération la démographie des territoires, afin que le déploiement de cette mesure réponde efficacement aux besoins de tous les Français, de manière égale, sur l'ensemble du territoire. L'accès aux psychologues ne devra pas être un frein à la bonne mise en oeuvre de ce dispositif important et nécessaire. Quel est l'avis de la commission ? L'article 42 prévoit déjà, dans son alinéa 9, que la répartition territoriale du nombre de psychologues pouvant proposer des séances d'accompagnement psychologique sera déterminée au regard des besoins de chaque territoire.

appuyée sur des conditions d'exercice représentatives, cet amendement vise à ne retenir que la participation de professionnels titulaires d'un minimum d'expérience professionnelle.

Ce protocole comprend des exercices ou travaux prescrits en vue de favoriser la rééducation ou le reclassement professionnel de la personne concernée. Eu égard aux dispositions présentes dans le décret, il semble nécessaire de renforcer la coordination et la coopération entre les acteurs et les différents protocoles, lors de la fin des traitements dans ces pathologies

le parcours de soins global après traitement d'un cancer a vocation à mobiliser des acteurs extrahospitaliers, notamment des partenaires associatifs, pour réaliser des bilans d'activité physique, ainsi que des consultations de suivi nutritionnel

L'amendement n° 326 rectifié apporte une coordination bienvenue dans le code de la sécurité sociale. Il vise à articuler le parcours de soins global post-traitement d'un cancer avec le protocole de soins que le médecin traitant doit élaborer pour les personnes atteintes d'une affection de longue durée

de prise en charge post-cancer. L'article 59 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 prévoit explicitement que le Gouvernement remettra au Parlement, d'ici à la fin de l'année 2021, un rapport dressant un bilan de ce forfait. Il n'y a donc

L'amendement vise à supprimer l'article 42. Le Gouvernement a été alerté depuis plusieurs années sur le problème du reste à charge des patients ayant recours à un transport sanitaire bariatrique. Pourtant, les solutions tardent à venir. Les négociations entre l'assurance maladie et les transporteurs sanitaires privés, qui devaient aboutir en 2021,

qui vise à demander la remise d'un rapport au Parlement sur la mise en oeuvre du parcours de soins global après le traitement d'un cancer, afin notamment d'étudier l'ouverture du remboursement des solutions thérapeutiques non hormonales favorisant le retour à une vie sexuelle normale des femmes après un cancer. Un tel rapport sur le forfait de prise en charge post-cancer est déjà prévu à l'article 59

S'agissant de l'amendement n° 383, un rapport de la Cour des comptes de 2018 pointe le reste à charge important des personnes présentant des troubles du spectre de l'autisme, non seulement sur les soins au sens strict, mais aussi sur les postes de dépenses comme les transports, les loisirs et séjours adaptés ou encore l'accompagnement à la guidance parentale. Cependant, conformément à la position de la commission sur les demandes de rapport, l'avis est défavorable.

Enfin, la reprise d'activité pour les personnes invalides est encouragée par un assouplissement réglementaire du cumul entre pension d'invalidité et revenu d'activité- c'était là encore un frein possible. On garantit

Si les implants mammaires et les prothèses mammaires externes sont pris en charge, les patientes ne peuvent être remboursées pour un tatouage tridimensionnel définitif de la plaque aréolo-mamelonnaire permettant une reconstruction esthétique du sein.

Les dispositions actuelles du code de la santé publique prévoient l'encadrement par décret des actes, procédés, techniques et méthodes à visée esthétique, car ils peuvent présenter des risques sérieux pour la santé des patientes.

Si ce modèle de réduction des risques a pu être critiqué par les tenants de la « guerre à la drogue », les études révèlent l'efficacité d'une approche globale et multiscalaire

Mme Raymonde Poncet Monge. Depuis leur ouverture en 2016 dans le cadre d'une expérimentation, les deux seules salles de consommation à moindre risque sont un succès que nous devons préserver et perpétuer. L'Inserm, qui est chargé de l'évaluation du dispositif, en rend compte dans son rapport remis en mai dernier.

Cet amendement vise à interdire l'implantation de haltes « soins addictions » à moins de 200 mètres des établissements et des services d'accueil de jeunes enfants, des établissements scolaires, des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et des infrastructures sportives.

est à Mme la rapporteure. L'expérience de la salle de consommation à moindre risque (SCMR) de Strasbourg montre les vertus d'un accueil des publics usagers de drogues dans des locaux situés aux abords des services hospitaliers. Cette proximité facilite la prise en charge des personnes les plus vulnérables qui peuvent présenter des pathologies justifiant une prise en charge médicale en urgence. En conséquence, cet amendement vise à privilégier la création des nouvelles haltes « soins addictions » dans l'enceinte d'établissements de santé- comme ce fut le cas

L'article 43, dans sa rédaction initiale, autorise l'ouverture de HSA soit dans les locaux du Caarud ou du Csapa, soit dans des locaux distincts. Il est donc possible de limiter leur ouverture à des locaux situés dans une emprise hospitalière ou à proximité immédiate.

à l'existence même de ces structures. La situation dramatique des jardins d'Éole, avec ses consommateurs de crack et, désormais, la construction d'un mur de la honte à Pantin, doit nous rappeler qu'il faut multiplier les structures d'accompagnement de soins plutôt que les obstacles à leur implantation.

le fonds de lutte contre les addictions permet de financer et d'amplifier des actions innovantes de prévention, d'accompagnement et de recherche sur les addictions liées à des substances psychoactives. Cependant, notre société évolue et les addictions d'hier ne sont pas forcément celles d'aujourd'hui. L'Inserm le souligne, la pratique des jeux de hasard, les paris sportifs, les jeux vidéo sont autant de pratiques qui peuvent avoir des répercussions médicales, psychologiques et psychiatriques sur le long terme.

du fonds de lutte contre les addictions en permettant qu'il finance des actions innovantes de prévention, notamment le soutien aux priorités du programme national de lutte contre le tabac et du plan national de mobilisation contre les addictions. Si nous souscrivons à cet objectif de santé publique, à savoir la promotion de la prévention des addictions, nous tenons à rappeler que le fonds de lutte contre les addictions n'est doté que d'une centaine de millions d'euros par an, soit 350 millions d'euros

de toutes les méthodes de contraception féminine, sur le remboursement des préservatifs féminins au même titre que les préservatifs masculins, ou bien encore sur la nécessité d'avancer concrètement à la gratuité de la contraception masculine, afin que cette question ne reste pas une charge mentale et financière supportée uniquement par les jeunes filles et les femmes.

C'est un fait, en 2021, on constate encore des inégalités dans l'accès à la contraception pour les femmes et les jeunes filles en particulier. Je me réjouis donc à mon tour que l'on puisse faciliter cet accès grâce à la gratuité et garantir encore un peu plus aux femmes le droit de disposer librement de leur corps.

mais je considère qu'il faudrait également étendre la mesure aux jeunes hommes de moins de 26 ans. Il s'agit d'une mesure de santé publique visant à limiter les risques de grossesse non désirée, ainsi que les risques de transmission des infections sexuellement transmissibles, en recrudescence chez les jeunes. La contraception n'est pas une responsabilité exclusivement féminine. Elle doit être partagée entre les femmes et les hommes. Je

les hommes bricolent, ils improvisent. Ce retard n'est plus possible. Nous avons collectivement trop tardé. Par cet amendement, nous demandons que le Gouvernement nous expose clairement pourquoi nous n'avançons pas suffisamment sur cette question et quel plan d'action il entend mettre en place pour rompre l'immobilisme des pouvoirs publics : immobilisme sur la recherche, sur la sensibilisation de la population, notamment des jeunes, sur la formation des professionnels de santé. Il est temps que la charge mentale de la contraception soit partagée, afin de lutter de manière concrète, notamment contre les rapports de domination au sein du couple. Au-delà des choix intimes qu'il revient à chacun

que ce rapport puisse être réalisé. Nous pensons utile que la Haute Autorité de santé puisse être associée à ces travaux pour contribuer à un état des lieux des connaissances et établir des recommandations sur l'ensemble

Mme Raymonde Poncet Monge. Encore aujourd'hui, les personnes trans sont exposées à des discriminations en raison de la rédaction « genrée » de la loi.

La jurisprudence du Conseil constitutionnel exige en effet que toutes les personnes placées dans des situations identiques soient soumises au même régime juridique et soient traitées de la même façon- sans privilège et sans discrimination. Tel est le principe constitutionnel que cet amendement tend à réaffirmer en garantissant l'accès des hommes trans de moins de 26 ans au remboursement de la contraception. Quel est l'avis

par rapport aux assurés femmes dans l'accès à la contraception gratuite. Quel est extrêmement attentif à ce que les personnes transgenres ne subissent aucune discrimination dans leur accès aux soins. Madame la rapporteure, le changement de mention du sexe à l'état civil ne fait pas obstacle à ce que les personnes transgenres puissent bénéficier de leurs droits, notamment en matière d'exonération de participation pour les frais liés à la contraception. Il ne paraît pas nécessaire d'inscrire cette doctrine dans la loi, car les caisses d'assurance maladie

entre les femmes et les hommes. La charge contraceptive, qu'elle soit mentale ou financière, pèse davantage sur les femmes. Il est vrai que celles-ci sont les premières concernées par la grossesse, donc les premières à devoir garantir leur droit à disposer librement de leur corps. Cependant, le coût de la contraception ne doit-il reposer que sur elles, nonobstant les méthodes contraceptives prises en charge par la sécurité sociale ? Cette injustice financière supplémentaire qui pèse sur les épaules des femmes n'est pas une fatalité. Cet amendement vise donc à demander au Gouvernement l'opportunité d'étudier la gratuité de toutes les contraceptions.

implant, dispositif intra-utérin, anneau, patch ... Les effets que l'on qualifie de secondaires ne le sont pas pour les femmes concernées. Au terme de ce parcours, le fait que la méthode contraceptive adaptée soit finalement payante- parfois très onéreuse - représente une injustice et une inégalité. Pour les femmes qui en ont les moyens, la contraception est une liberté ; pour les autres, c'est trop souvent la résignation qui l'emporte. Seule la contraception remboursée n'a pas de prix ; les effets secondaires, eux, pèsent au quotidien. Il s'agit donc de garantir un choix éclairé, accompagné bien sûr d'un avis médical, et libéré de toute pression financière. Quel est l'avis de la commission ? L'amendement

que seront concernés par la mesure de gratuité tous les produits contraceptifs pris en charge par l'assurance maladie, qu'il s'agisse des pilules de première et deuxième générations, des dispositifs intra-utérins, des implants, des diaphragmes ou des contraceptifs d'urgence.

féminins à hauteur de 60 %, comme les préservatifs masculins. Au contraire du préservatif masculin, largement promu et distribué, dont certains modèles sont remboursés sur ordonnance, le préservatif féminin, qui est méconnu, se vend à des tarifs entre trois à quinze fois plus élevés. S'il est vendu sans ordonnance dans certaines pharmacies, il demeure onéreux et difficile à trouver. Prévoir une possibilité de se faire prescrire ces préservatifs par les médecins et sages-femmes serait bénéfique.

Santé publique France publie d'ores et déjà régulièrement des baromètres santé qui fournissent des informations sur les pratiques contraceptives et les connaissances des Françaises et des Français sur le sujet. Cet amendement semble

Si l'on peut soutenir sur le fond les dispositions proposées, un tel article est déjà satisfait par le droit en vigueur, qui prévoit des examens postnataux obligatoires et relève, aux termes mêmes de la loi, du domaine réglementaire.

dans les premières semaines et les premiers mois qui suivent l'accouchement. L'article 44 , qui précise justement l'obligation de réaliser un entretien postnatal, est donc essentiel. Il l'est pour l'accompagnement des nouveaux parents, père et mère.

dans le pays. La fermeture des maternités porte à conséquence, car, toujours selon la Drees, près de 200 000 femmes en âge de procréer résident à plus de quarante-cinq minutes de la maternité la plus proche. Renforcer le maillage territorial et permettre à toutes les femmes d'être à proximité d'une maternité est donc un enjeu fondamental. À cet égard, le dispositif « engagement maternité avait justement pour objectif d'organiser des schémas territoriaux de prise en charge pour les parturientes qui résident à plus de quarante-cinq minutes d'une maternité. Il donnait également accès aux remboursements de prestations de transport ou à une prestation d'hébergement en hôtels hospitaliers, dont on connaît le faible développement. Il permettait aussi de définir dans chaque territoire les schémas d'accès aux soins de prévention, les prises en charge pré et post-partum, la permanence des soins périnataux et les mécanismes de prise en charge des urgences. En somme, il traçait des parcours lisibles pour les femmes. Pourquoi ce dispositif si essentiel reste-t-il encore limité à certains territoires ? Ce n'est pas entendable. C'est la raison pour laquelle l'amendement que nous présentons vise à demander une étude sur la faisabilité de l'extension de l'« engagement maternité » à l'ensemble du territoire et à prévoir son financement par une dotation populationnelle afin de répondre aux besoins des populations. Quel Nous avions ainsi voté en faveur d'une mesure facilitant l'accès aux soins pour les femmes enceintes les plus éloignées des maternités, grâce à une prestation d'hébergement temporaire non médicalisé ou à une prise en charge des frais de transport. Ces dispositions étaient toutefois insuffisantes pour pallier la désertification obstétricale engendrée par la fermeture des maternités : entre 1996 et 2016, le nombre de maternités a diminué de 39 % en France. Je souscris à votre intention d'améliorer l'accès aux maternités sur le territoire.

dise, et la complexité technique du sujet ont retardé la publication des textes d'application. En particulier, la définition du critère des quarante-cinq minutes a nécessité- croyez-moi sur parole -d'importants travaux de la Drees. Ces Ces travaux sont achevés et des projets de textes viennent d'être soumis au ministre des solidarités et de la santé. Nous nous engageons à ce qu'ils soient publiés très rapidement, d'ici à la fin de l'année.

mais sérieusement, monsieur le ministre, après des mois de mobilisation de ces professionnelles pour faire reconnaître davantage leur profession, n'avez-vous rien d'autre à leur proposer qu'une campagne de communication ? Je ne suis pas certaine

de sage-femme ! Sinon, comment expliquer que, face au mouvement de contestation mené le mois dernier par les sages-femmes, rien ou presque n'ait bougé ? Une prime exceptionnelle de 100 euros a été prévue, ainsi qu'une hausse de salaire. Ce n'est pas négligeable, mais vous voyez bien que ce n'est pas suffisant pour redonner de l'attractivité à ce métier et pour le reconnaître à sa juste valeur. Lors de la grève, je vous rappelle que, sur les 500 maternités de France, 150 comptaient 100 % de grévistes. Le mouvement a également été très suivi chez les sages-femmes libérales, avec 60 % des cabinets fermés. Ce qu'elles demandent, ce n'est pas une campagne d'information, mais c'est notamment d'obtenir le statut de

qui vient, hélas, de nous quitter, et qui était très engagé sur cette question comme sur la défense de l'IVG ou encore des hôpitaux et des maternités, et plus largement de la médecine de proximité. Un statut de praticien médical permettrait par exemple aux sages-femmes de faire de la recherche en parallèle,

pour lesquelles les membres de la commission des affaires sociales ont beaucoup de respect, méritent mieux qu'un article introduit par voie d'amendement dans ce projet de loi de financement de la sécurité sociale

de faire une campagne de promotion des compétences des sages-femmes, qui ont beaucoup évolué ces dernières années et qui sont assez peu connues du grand public, constitue une

pas vous laisser dire, madame Cohen, que notre action et notre engagement en faveur des sages-femmes se limitent à une campagne de communication, car ce n'est pas vrai. Il y a eu, effectivement, une revalorisation de 183 euros, dans le cadre du Ségur de la santé. Il y a eu la prime de 100 euros.

Le présent article prévoit que la première consultation, pour une demande de stérilisation à visée contraceptive, puisse se faire auprès d'une sage-femme et non plus seulement auprès d'un médecin. médecin. Il concerne les missions des professionnels de santé, mais n'a pas d'incidence sur l'équilibre financier des régimes de sécurité sociale. Il ne relève donc pas du domaine des lois de financement de la sécurité sociale.

Nous sommes défavorables aux amendements de suppression de cet article, qui permet une forme d'expérimentation, puisque les sages-femmes pourront réaliser la première consultation d'information auprès de femmes qui feraient une demande de stérilisation à visée contraceptive.

foyer. Très concrètement, il vous est d'abord proposé d'ouvrir le contentieux aux décisions relatives aux organismes complémentaires, ce qui va permettre une mise en cohérence du champ du contentieux relatif à ce dispositif. un peu technique, mais importante ... En outre, il vous est proposé d'ajouter les réductions de dettes et les aides accordées par les organismes complémentaires aux situations pour lesquelles un assuré pourra tout de même se voir attribuer un droit à la complémentaire santé solidaire s'il ne s'est pas acquitté de l'ensemble de ses participations financières. Cela vise à éviter au maximum les ruptures de droits, tant que l'assuré est de bonne foi. Enfin, il est prévu des exceptions à la durée d'un an du droit à la complémentaire santé solidaire, afin de résoudre les problèmes qui nous ont souvent été signalés par les associations. En effet, en cas d'arrivée d'une nouvelle personne dans un foyer bénéficiaire de la complémentaire santé solidaire, cette personne devait attendre l'expiration du droit du foyer pour bénéficier de la C2S. Cette mesure permettra de permettra de donner plus de souplesse aux assurés pour pouvoir s'adapter à l'évolution de leur situation familiale, et contribuera ainsi à réduire les renoncements aux soins - c'est bien de cela dont il s'agit,- en facilitant l'accès à la complémentaire santé solidaire. Quel est l'avis de la commission ? Cet amendement

à combler un vide juridique en élargissant le contentieux d'admission à l'aide sociale aux décisions prises vis-à-vis des organismes complémentaires. Il vise à étendre la possibilité de renouveler le droit à la C2S, même si l'assuré ne s'est pas acquitté de sa participation financière, au cas où il fait l'objet d'une réduction de dette. La commission est favorable à ces évolutions. Par ailleurs, l'amendement prévoit des exceptions à la durée d'un an du droit à la C2S. Si elles sont favorables aux bénéficiaires, ces dispositions devraient donner lieu à des difficultés de gestion très importantes pour les services compétents.

disposition - ce qui est une avancée à saluer - et que les personnes en situation de handicap en soient exclues, alors qu'elles sont exposées, elles aussi, à de forts restes à charge liés à des dépenses de soins plus élevées.

sont un public particulièrement précaire et présentent un taux élevé d'absence de couverture par une complémentaire santé, alors même qu'une partie d'entre eux pourrait avoir droit à la complémentaire santé solidaire. Cet amendement vise donc à offrir une égalité de traitement entre les bénéficiaires de l'AAH et ceux de l'ASPA.

les bénéficiaires de l'AAH et de l'ASI, sous les mêmes conditions, à savoir l'absence d'activité professionnelle. En effet, la grande majorité de ces bénéficiaires sont éligibles à la complémentaire santé solidaire.

affection de longue durée non déclarées, mais connues de l'assurance maladie. Enfin, les informations complémentaires potentiellement nécessaires pourraient être sollicitées auprès des bénéficiaires. Cette mesure permettrait de faciliter le maintien de la couverture complémentaire pour des personnes susceptibles d'avoir des besoins de santé importants.

L'accès la C2S avec participation est conditionné à la perception de revenus compris entre 753 euros et 1 017 euros. C'est notamment la raison pour laquelle, avec cet article 45, les allocataires de l'ASPA, dont le montant est fixé à 907 euros, seraient réputés remplir les conditions d'ouverture du droit à la complémentaire santé solidaire

leurs allocataires, lorsqu'ils n'exercent pas d'activité professionnelle, doivent également pouvoir accéder facilement à la complémentaire santé solidaire avec participation. Le bénéfice de cette C2S est de nature à améliorer les conditions d'accès aux soins des personnes les plus précaires.

période au cours de laquelle sont étudiées les ressources n'est pas identique : année pour l'AAH contre les douze derniers mois glissants pour la C2S. Les ressources que l'on prend en considération ne sont pas non plus comparables, celles étudiées pour la C2S étant plus larges.

les personnes en situation de handicap, se trouvent en grande précarité. Chaque année, nous décidons de mesures d'accompagnement pour elles, mais force est d'admettre que, comme de nombreuses études le signalent, le taux de non-recours aux aides sociales se situe autour de 40 %.

C'est la raison pour laquelle nous vous proposons d'inverser le principe de l'allocation de la complémentaire santé solidaire en confiant à l'organisme verseur la charge d'étudier l'éligibilité des allocataires. La parole

complémentaire santé. Lutter contre le non-recours aux droits et prestations implique d'aller au-delà des campagnes d'information et d'expérimenter l'attribution automatique de la C2S à l'ensemble des bénéficiaires de minima sociaux, comme le recommandent plusieurs rapports récents, dont celui de la Cour des comptes en juin 2021. Nous proposons donc, par cet amendement, un premier pas vers l'automatisation des droits, en mettant en oeuvre une étude systématique de l'éligibilité à la C2S, qui s'appuiera sur les ressources connues par les différentes administrations. Par ailleurs, cet amendement vise à prévoir une information des modalités d'accompagnement en vue de la résolution de la situation de l'assuré n'ayant pu s'acquitter de l'ensemble de ses cotisations, afin de ne pas pénaliser ceux qui, en difficulté financière,

Toutefois, les derniers chiffres de l'assurance maladie montrent un taux élevé de non-recours de ces bénéficiaires à une complémentaire santé. Ce constat a également été dressé par la Cour des comptes dans son rapport de juin 2021 intitulé Parmi ses Parmi ses recommandations, la Cour invite le législateur à s'engager rapidement vers l'attribution automatique de la C2S à l'ensemble des bénéficiaires de minima sociaux. Si cette ambition peut se heurter au manque d'interopérabilité des systèmes d'information et des bases de données des différents organismes sociaux, l'obstacle n'est pas infranchissable. preuve, l'attribution automatique de la C2S aux bénéficiaires du RSA a longtemps été refusée pour ces raisons avant d'être finalement mise en oeuvre dans le cadre de cet article. Le présent amendement vise donc à développer cette ambition d'attribution automatique en s'appuyant sur les ressources déjà connues par les différents organismes sociaux CAF, MSA et CNAM. Il s'agit de poursuivre le processus de lutte contre le non-recours aux droits et prestations engagé depuis 2017 et de permettre l'accès à une couverture complémentaire aux plus fragiles de nos concitoyens. La parole est à Mme Monique Lubin,

Lubin. Cet amendement vise à mieux informer les assurés des modalités d'accompagnement pour recouvrer leurs droits. En effet, le potentiel bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé peut se voir refuser le renouvellement de son droit s'il ne s'est pas acquitté d'une seule mensualité. Nous proposons donc qu'il soit informé des modalités d'accompagnement pour résoudre sa situation par une action sanitaire et sociale pour le paiement des des cotisations dues, afin de permettre la réouverture de ses droits. Nous souhaitons évidemment, comme vous tous- j'imagine -, que l'accompagnement soit privilégié pour éviter les ruptures de droits et de parcours de soins. Mme Raymonde Poncet Monge. À ce jour, on estime que près de la moitié des personnes sans couverture santé complémentaire pourraient prétendre à la complémentaire santé solidarité.

sur les modalités d'accompagnement pour permettre la réouverture ou le renouvellement du droit à la C2S. D'abord, une telle mesure entraînerait une charge supplémentaire pour les services concernés. Surtout, l'article prévoit déjà une aide au paiement des participations par les caisses d'assurance maladie ou les organismes complémentaires. Celle-ci permet justement aux bénéficiaires d'assurer

du dispositif jusqu'à la veille du vingt-quatrième anniversaire. Le régime local couvrant les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est un régime autonome de sécurité sociale. Le rehaussement s'alignera avec les dispositions de droit commun, à savoir l'âge fixé pour l'affiliation au régime d'assurance maladie des parents pour les enfants sans activité professionnelle, en application de la loi du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants.

Cette gestion comprend le contrôle des prescriptions, de la délivrance et le remboursement des frais d'optique pour la part du régime obligatoire et la part du régime complémentaire.

tout en permettant à l'assurance maladie de conserver la récupération des données de prescription, de délivrance et de remboursement, ainsi qu'un contrôle de l'ensemble des opérations réalisées par les complémentaires, la production de rapports annuels exhaustifs présentant une vision globale de l'évolution des dépenses. Quel est l'avis de la commission ? Cet amendement vise du panier de classe B, pour lequel les prix sont libres, par opposition à la classe A, constitutive du panier « 100 % Santé », pour laquelle les restes à charge sont nuls. Si la commission ne s'y oppose pas par principe, elle estime nécessaire de travailler préalablement le sujet plus en profondeur, en associant les complémentaires santé, les organismes d'assurance maladie et les professionnels. La question est donc sur la table et elle doit être débattue. En attendant, je demande le retrait de cet amendement

Le bénéfice du tiers payant intégral est indispensable pour permettre un accès pleinement effectif aux équipements du panier « 100 % Santé ». C'est une condition de réussite essentielle de la réforme, compte tenu des montants importants que peut représenter l'avance de certains soins de dispositifs médicaux pour les personnes.

la simplification des outils mis à disposition permettra aux professionnels d'accroître le recours au tiers payant intégral, donc d'améliorer l'accès aux soins de tous les assurés. C'est la raison pour laquelle il nous semble opportun de mettre en place une telle mesure sans attendre. Son inscription en loi de financement de la sécurité sociale

et prestations sociales. Nous proposons de faire de l'échange des données entre les différentes administrations un outil d'attribution des droits sociaux, et non simplement d'information des usagers sur les mécanismes auxquels ils ont droit.

Quel est l'avis de la commission ?

Le présent amendement vise à actualiser un état des lieux peu encourageant de l'accès aux soins des plus précaires dans notre pays. À la suite d'une enquête menée conjointement avec le fonds 2019 auprès de 1 500 cabinets médicaux de gynécologues, chirurgiens-dentistes et psychiatres, le Défenseur des droits a révélé que 10 % des praticiens ont été pris à refuser des soins aux patients bénéficiant de la CMU-C ou de l'ACS. Il ne s'agit là toutefois que d'une moyenne nationale. Les refus de soins discriminatoires sont très variables selon les régions, ce qui n'avait pas pu être montré jusqu'ici, souligne le rapport. À Paris, ce sont près de quatre dentistes sur dix, d'un gynécologue sur quatre et d'un psychiatre sur trois qui refusent des patients en situation de précarité économique. Les auteurs de l'étude qualifient ces refus de soins de « discriminatoires, explicites et directs ». Si le code de la santé publique prévoit effectivement qu'un médecin puisse se dégager de sa mission de soins pour des raisons professionnelles ou personnelles tout en garantissant la continuité des soins à ses patients ou en orientant ceux qu'il ne peut prendre en charge vers un de ses confrères, l'article L. 1110-3 du même code interdit formellement le refus de l'accès aux soins d'une personne

et la nature des pratiques de refus de soins par les moyens qu'ils jugent appropriés ». Une commission d'évaluation des pratiques de refus de soins a été mise en place auprès du conseil national de l'ordre des médecins. Le rapport qu'elle a remis au Gouvernement au mois d'octobre 2020, 2020, couvrant la période de juillet 2019 à juillet 2020, dresse le constat d'une « situation peu ou pas évaluée dans sa globalité par manque de moyens ». La publication par le Gouvernement du décret du 2 octobre 2020 relatif à la procédure applicable aux refus de soins discriminatoires et aux dépassements d'honoraires abusifs ou illégaux, appliqué depuis le mois de janvier 2021, peut constituer un début de réponse.

45 vise à codifier des dispositions nouvelles relatives au dispositif mis en place par l'article L. 160-3 du code de sécurité sociale. La proposition de la commission comporte, selon nous, des inconvénients. En effet, il n'est pas d'usage de codifier des dispositions non pérennes. Or la rédaction envisagée concerne un nombre limité de personnes et couvre des situations ayant vocation à disparaître avec le temps. Dans un souci de clarté des dispositifs en vigueur, le code de la sécurité sociale ne peut comporter que des mesures pérennes et de portée générale. Il nous semble donc plus adapté de prévoir une bonne information des retraités expatriés qui bénéficient de ce droit au 1 juillet 2019, relayée par les organismes de sécurité sociale et leurs élus.

sous peine d'incompatibilité avec une prise de décision médicale. Il s'agit d'éviter ainsi l'engorgement actuel des rendez-vous médicaux physiques, dans un souci de justice sociale et d'efficacité.

effectivement exister un problème d'accès au second avis pour les personnes souffrant d'une pathologie grave. La commission partage ce constat. Toutefois, la vidéotransmission entraîne déjà une forte perte d'informations pour le médecin.

Par ailleurs, le traitement d'une pathologie lourde mérite mieux qu'un entretien téléphonique. S'il peut exister un problème d'accès au second avis, le véritable sujet à traiter serait celui de l'accessibilité directe et physique au médecin. La solution pourrait résider dans une meilleure prise en charge de transport pour ces patients plutôt que dans le soutien

Or ils subissent des différentiels de traitement inadmissibles et injustes. Il est impératif de réformer notre système social, afin qu'il ne soit plus pénalisant pour nos concitoyens Les travailleurs les plus précaires, qui ont les carrières les plus courtes et les plus hachées- ce sont souvent des femmes qui accompagnent leur compagnon à l'étranger -, subissent les règles de calcul des retraites actuelles. Par exemple, la décote est une véritable double peine pour les carrières et son effet est amplifié par la situation des Français de l'étranger. Certains retraités sont confrontés, par exemple au Liban ou au Venezuela, à des situations absolument catastrophiques

! Quel est l'avis de la commission ?

parole est à Mme la rapporteure. Cet article prévoyait à l'origine la possibilité de prendre jusqu'au 31 décembre 2022 des mesures dérogatoires, non seulement en matière de prise en charge des frais de santé et de bénéfice des prestations en espèces, mais également d'indemnités L'Assemblée nationale a procédé, par amendement du Gouvernement, au retrait des dispositions relatives aux indemnités complémentaires pour les introduire dans le projet de loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, à son article 5 , mais en remplaçant l'échéance du 31 décembre 2022 par celle du 31 juillet 2022. Il est dès lors permis de se demander pourquoi cette date était fixée au 31 décembre dans le PLFSS originel s'il est finalement possible de l'avancer et ce, d'autant plus que les mesures dérogatoires déjà prises dans ces domaines en 2021 ont représenté pour l'assurance maladie un coût élevé en 2020-

relatives au versement de l'indemnité complémentaire pouvaient être maintenues. En cohérence avec cette position, la commission propose d'avancer du 31 décembre 2022 au 28 février 2022 l'échéance jusqu'à laquelle, d'une part, le délai de carence applicable aux agents publics et à certains salariés serait suspendu et, d'autre part, des mesures dérogatoires en matière de frais de santé et de bénéfice des prestations en espèces pourraient être maintenues.

prises par décret et relatives à la prise en charge des frais de santé et au bénéfice des prestations en espèces. Les dispositions contenues dans les ordonnances en question ne seraient applicables que jusqu'au 31 décembre 2022 et chaque ordonnance pourrait prévoir l'application rétroactive des dispositions qu'elle contient jusqu'à un mois avant la date de sa publication. Cette habilitation ne se justifie pas, au regard de l'ampleur des mesures dérogatoires au droit commun, et donc à la loi, déjà prises en 2020 et 2021 sans une telle habilitation. Le champ des dérogations à la loi est déjà suffisamment large sans qu'il soit besoin d'empiéter encore davantage sur la compétence du législateur grâce à un champ d'habilitation démesurément vaste. En effet, les ordonnances relèveraient de dispositions relatives à la prise en charge des frais de santé et au bénéfice des prestations en espèces, en présence d'un risque sanitaire grave et exceptionnel, et ne seraient pas directement en lien avec le risque en cause, mais nécessaires à la limitation des effets de ce risque. Par ailleurs, la commission a préconisé de supprimer la même habilitation en matière d'indemnités complémentaires figurant dans le projet de loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, étant donné le flou absolu sur les intentions du Gouvernement que l'on retrouve dans la formulation de cet article.

Cet article prévoit la reconduction, y compris par ordonnances, des mesures visant à faire face à la covid-19, notamment la prise en charge renforcée des frais de santé, l'amélioration des conditions d'accès aux soins et le versement de certaines indemnités. Il prévoit notamment de prolonger la suppression du jour de carence en cas de congé maladie directement lié à la covid-19, pour certains agents publics et salariés. Le rapport pour avis sur le projet de loi de Marche, Émilie Chalas, consacré à la fonction publique, indique que le rétablissement du jour de carence dans la fonction publique a eu, sur l'absentéisme, un résultat mitigé en dehors de la période de pandémie. En outre, durant la crise sanitaire, il n'y a pas eu d'explosion du nombre de congés maladie dans la fonction publique. Cela tend à prouver, si besoin était, que les jours de carence n'ont qu'un effet à la marge sur le comportement des agents du service public. Nous sommes opposés, vous le savez, à ces jours de carence et nous espérons que le prochain gouvernement aura le courage de tirer les conclusions qui s'imposent, en supprimant ce délai pour les salariés et les fonctionnaires. Je mets aux voix

est à Mme la rapporteure. Cet article permet à Santé publique France de céder à titre gratuit ses biens meubles, tels que les masques et dispositifs médicaux divers, à des organismes publics, afin d'en assurer le renouvellement ou d'en éviter la destruction.

déduire des éventuelles économies réalisées par Santé publique France une diminution concomitante de cette dotation. Ainsi, et de position constante, la commission estime que cette mesure est irrecevable au titre de l'article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale. La commission vous demande donc de procéder à sa suppression.

effet, elle contribuera à optimiser les dépenses d'un opérateur financé par l'assurance maladie. Je rappelle, d'ailleurs qu'elle sera également favorable aux établissements de santé et, au-delà, à de nombreux organismes chargés d'une mission de service public, puisqu'elle leur permettra de réduire leurs dépenses d'achat à concurrence des cessions que Santé publique France réalisera à leur profit.

parole est à Mme la rapporteure. Le présent article vise à permettre de nouvelles transmissions de données de santé, notamment aux praticiens de santé ou dans le cas de menaces sanitaires. Si l'intention est louable, le dispositif relève d'une loi de santé et ne répond pas au champ des lois de financement de la sécurité sociale défini par la loi organique.

territoires. Il a pour objet la mise en place d'un capital décès, destiné à apporter un soutien financier aux familles des non-salariés agricoles, lorsqu'elles sont confrontées au décès d'un des leurs après une maladie, un accident de la vie privée ou un suicide. Contrairement aux autres régimes de sécurité sociale, le régime des exploitants agricoles ne prévoit pas l'attribution d'un capital décès aux ayants droit survivants, qu'il s'agisse du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, des enfants ou des ascendants. La mesure proposée vise donc à corriger cette différence de couverture sociale, dans une démarche d'harmonisation et de renforcement de la protection des exploitants agricoles. Elle répond à un engagement du plan gouvernemental d'accompagnement des agriculteurs en détresse et de prévention du suicide, en permettant à la Mutualité sociale agricole (MSA) d'améliorer l'aide apportée aux familles en cas de suicide du chef d'exploitation ou d'un membre de la famille travaillant sur l'exploitation. Le montant du capital décès qu'il est proposé d'attribuer aux familles des non-salariés agricoles décédés en activité est équivalent, par équité entre assurés agricoles, agricoles, à celui garanti aux ayants droit des salariés agricoles, soit un montant forfaitaire de 3 476 euros en 2021. Sur le plan financier, l'instauration de ce capital décès se traduira par une charge estimée à 2,9 millions d'euros pour le régime maladie-maternité-invalidité des exploitants agricoles (Amexa), qui sera financée sans aucune augmentation de la cotisation.

commission est favorable sur ces trois amendements, qui mettent fin à une différence de traitement difficilement explicable entre les non-salariés agricoles et les autres régimes de sécurité sociale, au désavantage des premiers. La possibilité qui est ouverte à leurs ayants droit de percevoir un capital décès va dans le sens d'une plus grande équité.